d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale

! C’est tout le sens de l’agenda que le Premier ministre a défini pour ce gouvernement. La France, quant à elle, a de solides arguments à faire valoir. L’activité se maintient : le taux de croissance pour 2024

Ce niveau de dette affecte notre souveraineté, notre crédibilité et notre capacité à aborder l’avenir de manière concrète : nous paierons bientôt plus de 50 milliards d’euros d’intérêts par an.

Mesdames, messieurs les sénateurs, on trouve toujours des justifications pour augmenter les dépenses. Ce n’est jamais le bon moment pour faire des économies… Il est toujours tentant de laisser le problème à ses successeurs. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins.

de notre pays et donc de renforcement de notre souveraineté financière nationale. J’insiste sur le fait que cet objectif doit être atteint priorité par des baisses de dépenses. Notre dépense publique étant devenue la plus importante de l’Union européenne, sa réduction constitue l’essentiel de l’effort qui vous est aujourd’hui proposé. Il nous faut maîtriser la dépense et l’emploi public, simplifier le fonctionnement de l’État, réduire son train de vie et

vous avez eu l’occasion de débattre en commission des finances, ont été conçus pour affecter le moins possible la croissance et pour poursuivre la décarbonation de notre économie.

ai je besoin de le répéter ? – que ces prélèvements soient exceptionnels, temporaires et ciblés. Nous proposons également de décaler la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui était initialement prévue.

Mesdames, messieurs les sénateurs, chacun devra contribuer – l’État, les collectivités locales, la sphère sociale –, non pas parce qu’il existerait de bons et de mauvais gestionnaires, certains qui dépensent bien et les autres, mais parce que l’effort à fournir nécessite l’engagement de tous. la réduction du train de vie de l’État est une condition indispensable pour justifier des prélèvements supplémentaires, même si elle est parfois symbolique, nos compatriotes étant attentifs aux efforts que nous sommes capables de faire. Elle est aussi une condition indispensable pour justifier des prélèvements supplémentaires afin de ramener le déficit

Dans le contexte politique que nous connaissons, et après le rejet du projet de budget par l’Assemblée nationale, le Sénat a plus que jamais une responsabilité majeure ; je ne doute pas que chacun d’entre vous en ait conscience.

Nos priorités économiques sont claires : réindustrialiser le pays et atteindre le plein emploi. Vous connaissez les réformes qui ont été menées à cet effet. Je pense à la baisse de la fiscalité pesant sur les entreprises, à la baisse des impôts de production, ou encore à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

la responsabilité budgétaire collective à laquelle nous appelons implique un plus grand souci de transparence et d’exactitude. La situation actuelle exige un renforcement du pilotage de nos finances publiques et une plus grande association de la représentation nationale.

de la dépense publique. Nous avons ainsi installé un comité scientifique, qui rendra des préconisations techniques pour améliorer nos prévisions dans ce nouveau contexte

je me réjouis d’entamer avec vous aujourd’hui l’examen du projet de loi de finances pour 2025. Comme vous le savez, conformément à notre Constitution, le rejet de la première partie du texte

logement. À cet égard, plusieurs propositions intéressantes émanent de vos travées, dont certaines rejoignent des initiatives dont nous avons débattu à l’Assemblée nationale ; les échanges que nous avons eus en commission l’ont bien démontré.

Nous pourrons améliorer ce projet de budget pourvu que le cadre de responsabilité fixé par le Gouvernement soit respecté. Vous le savez, le texte initial du Gouvernement suit une ligne de crête entre, d’un côté, l’exigence de protéger le pouvoir d’achat des Français les fondamentaux de notre économie et, de l’autre, la nécessité de renouer avec une trajectoire des finances publiques soutenable. Concrètement, il s’agit d’engager immédiatement un effort de redressement inédit de nos finances

Notre horizon doit rester celui de la prévisibilité fiscale. C’est la condition d’une politique économique efficace. Nous l’avons inscrit clairement dans le texte, qu’il s’agisse des contributions exceptionnelles sur les ménages ou sur les entreprises. Dans un pays où

prennent à leur charge la moitié des économies nécessaires, soit plus de 21,5 milliards d’euros. Comme je l’avais annoncé devant votre commission des finances, nous avons, faute de temps,

de l’attractivité, tout en redressant nos comptes publics. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission, mes chers collègues,

Évidemment, les contingences de notre vie politique l’expliquent largement. Mais le contexte économique et budgétaire dans lequel nous sommes amenés à nous prononcer l’explique tout autant, car il est à l’origine du contenu même du projet

recul. Faute de comprendre la situation économique et budgétaire de notre pays, on ne peut pas comprendre ce budget, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le voter. La France vit certes à crédit depuis cinquante puisqu’elle est en déficit depuis 1975, mais le déficit annuel et la dette, qui s’accumule, ne sont pas en soi un problème, loin de là. Ils nous permettent en effet de préparer l’avenir et de gouverner la France dans le temps long, celui de notre horizon commun. Cela reste vrai tant que deux limites ne sont pas franchies : celle qui établit, chaque année, que le remboursement de cette dette reste soutenable, et celle qui traduit le fait que les investisseurs veulent bien nous prêter, et dans de bonnes conditions. La règle des 3 % de déficit est certes conventionnelle, mais force est de constater qu’elle est très protectrice, car elle permet, peu ou prou, d’éviter ces deux écueils. Or que s’est il passé depuis 2022 ? En 2022, le déficit public de notre pays était déjà très élevé, puisqu’il s’élevait à 4,8 % du PIB. En 2023, alors que tous nos partenaires européens, soumis au même contexte économique, réduisaient fortement leur déficit, la France, elle, laissait ses comptes se dégrader sérieusement de 4,8 % de déficit, nous passions à 5,5 %, et ce sans récession, sans choc, sans raison particulière. Malheureusement, ce déficit n’est resté historique qu’un an : dès cette année, il est prévu atteigne 6,1 % du PIB, toujours sans récession, sans choc, sans raison particulière. Et ce qui devait arriver arriva. D’une part, la charge de la dette, mot convenu pour désigner en réalité ce que les Français doivent rembourser chaque année,

ces 70 milliards d’euros supplémentaires sont soit de l’impôt en plus, soit des dépenses en moins ailleurs. D’autre part, les conditions d’emprunt se dégradent : la France emprunte désormais plus cher que l’Espagne, le Portugal ou la Grèce, pays dont je rappelle qu’il frôlait la cessation de paiements il y a dix ans.

aussi un regret : de ces 50 milliards d’euros d’écart, personne n’endosse la responsabilité. Tous les responsables politiques que nous avons auditionnés ont répondu d’une même voix qu’ils n’étaient responsables de rien, ou de si peu,

« C’est pas moi », « c’est pas ma faute », « pas de bol ! » : comment lutter contre la crise démocratique quand les responsables politiques n’assument même pas la trajectoire des finances publiques du pays qu’ils dirigent ?

Mettons fin à cette mystification : il est temps de dire la vérité aux Français. J’approuve ce budget pour ce qu’il est : un budget de vérité,

L’année dernière, les dépenses de l’État continuaient d’augmenter, encore et encore, de près de 6 milliards d’euros, hors mesures de crise, par rapport à 2023. Au total, retraitées de l’inflation, les dépenses de l’État ont ainsi progressé de 14 soit une hausse historique. Je me réjouis que ce projet de loi de finances signe, enfin, la fin du « quoi qu’il en coûte ». Il aura fallu quatre ans pour nous désintoxiquer de la dépense publique. Pour 2025, le Gouvernement prévoit « enfin », oserais je dire, que les dépenses de l’État baissent de 3,2 %. L’effort, qui n’est pas lié au retrait des mesures de crise,

La voie est donc claire : il nous faut réduire la dépense publique. La commission des finances proposera d’aller plus loin en ce sens, non pas par dogmatisme, mais pour nous permettre de sortir du marasme budgétaire, tout en évitant au maximum des hausses d’impôts qui pèseraient sur les Français.

J’entends bien sûr les remarques, qui émanent de certaines travées, sur la nécessité de réformes structurelles pour faire baisser la dépense. Autant vous le dire, je les partage, nous les partageons ! Mais, je le rappelle, le Gouvernement a été nommé le 21 septembre 2024

À court terme, notre priorité est et doit être de préserver le pouvoir d’achat des Français, et non de préserver telle ou telle enveloppe budgétaire ou tel ou tel opérateur. Pour ce faire, il faut faire des économies et éviter les hausses de fiscalité. C’est cet objectif qui a guidé notre commission des finances dans son refus de la proposition gouvernementale d’augmentation de la fiscalité sur l’électricité au delà de son niveau d’avant crise. le prix de l’électricité va baisser, messieurs les ministres ! Oui, c’est une bonne nouvelle pour les Français ! Et, ne vous en déplaise, cela ne doit pas être l’occasion pour l’État d’augmenter subrepticement les impôts ! La commission des finances du Sénat propose 3,4 milliards d’euros d’impôts en moins et, donc, de pouvoir d’achat en plus pour les Français. Messieurs les ministres, vous êtes ici dans la maison des collectivités territoriales. Le rôle constitutionnel du Sénat est bien sûr de les représenter.

C’est l’État qui emprunte pour payer ses dépenses de fonctionnement courant. C’est donc l’État qui doit faire l’essentiel de l’effort de redressement de nos comptes publics. Aussi, je me réjouis

Par ailleurs, comme je l’ai déjà indiqué à de nombreuses reprises, y compris à cette tribune, je suis favorable à un effort des collectivités locales pour redresser nos comptes publics. Je rappelle que nous sommes dans une

Je suis sûr, messieurs les ministres, que vous n’êtes pas dupes : vous savez que sous le joli mot d’« arbitrage de dividendes » se dissimulent des pratiques organisées de démarchage de clients dans le but exclusif de frauder l’impôt.

Certes, dans un monde idéal, le gouvernement de Michel Barnier ne serait pas arrivé au pouvoir dans un contexte où le déficit public risquait d’atteindre 7 % du PIB.

Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en ma qualité de président de la commission des finances, et alors que s’engage l’examen du projet de loi de finances pour 2025, je débuterai mon intervention en rappelant que cela fait plus d’un mois déjà que le rapporteur général et l’ensemble des rapporteurs spéciaux procèdent à l’analyse de ce nouveau budget, tant de son volet recettes que de son volet dépenses. Je remercie l’ensemble des membres de la commission, ainsi que les rapporteurs pour avis, de la qualité de leurs travaux et des échanges qui ont nourri nos réunions.

celui de proposer un texte qui pourrait être la base des discussions lors d’une future commission mixte paritaire, nous ne pouvons que collectivement regretter que le texte initial du Gouvernement n’ait pas été complété par les propositions de l’assemblée la plus représentative de l’état le plus actuel de l’opinion, et que le volet dépenses n’ait même pas été examiné.

réduire significativement notre niveau de déficit pour diminuer notre appel à l’emprunt, et tout cela sans peser ni sur la qualité de nos services publics ni trop fortement sur une croissance que l’état de notre économie, comme celui de l’environnement international, ne nous permet guère d’imaginer très élevée. élevée. Notre débat portera donc sur les voies et moyens d’y parvenir. Or, comme toujours, le diable se cache dans les détails des mesures proposées. Au moins n’entendons nous plus dire que l’augmentation des impôts serait une ligne rouge par ceux là mêmes qui, pourtant, sont responsables de la situation actuelle. Quelles qu’aient pu être les motivations des baisses d’impôts décidées depuis 2018 et qu’elles aient été partagées ou non, lesdites baisses auraient dû être stoppées dès le début de la crise du covid

pour plus de 5 milliards d’euros à ce jour et 8 milliards d’euros au total programmés d’ici à 2029, selon votre texte, messieurs les ministres. Nonobstant les crises violentes et la nécessité de mesures de soutien exceptionnelles, mises en œuvre

! … bien plus permanent pour les ménages et les collectivités locales. Avant d’aller plus loin et de débattre des articles de ce projet de loi de finances, il ne serait peut être pas inutile de porter un jugement sur cette politique de baisse des recettes fiscales. Pour ce qui est de la taxe d’habitation, la mesure initiale de suppression de l’impôt pour 80 % des ménages a coûté 9 milliards d’euros. Son extension

qui s’était stabilisé à 12,9 % au premier trimestre 2018, a grimpé à 17,6 % au deuxième trimestre 2024, l’un des taux d’épargne les plus élevés d’Europe.

l’État aura rendu aux plus aisés ce qu’il propose maintenant de prélever sur tous : une sorte de « Robin des bois », mais à l’envers Le même raisonnement vaut pour les impôts de production : il a été impossible à France Stratégie, organe placé auprès du Premier ministre, d’évaluer l’impact de la suppression, pour 15 milliards d’euros à ce jour, de différents impôts de production.

non gagées par ses prédécesseurs. Avec une surtaxe sur deux ans des très grandes entreprises, il revient de fait, certes temporairement, sur la baisse de 33 % à 25

Le Gouvernement considère d’ailleurs, comme vous le savez, que la suppression d’exonérations de cotisations patronales est une baisse de la dépense et non une augmentation des recettes. Aussi ma proposition consiste t elle

Mes chers collègues, la crise des finances publiques que nous connaissons doit nous permettre de revenir sur nos erreurs. Ne laissons pas passer cette chance unique,

si quelqu’un a quelque raison que ce soit de s’opposer à ce mariage, qu’il parle maintenant ou se taise à jamais Si vous êtes favorables, mes chers collègues, au rétablissement d’un pouvoir fiscal pour les collectivités locales, dites le aujourd’hui en votant mes amendements, ou alors n’en parlez plus jamais !

Notre groupe n’a jamais refusé de débattre, bien au contraire. La question n’est donc pas celle du débat en lui même, mais de ce sur quoi il nous est demandé de débattre aujourd’hui. Ce projet de loi de

La gauche a ainsi démontré qu’un autre budget pour la France était possible : un budget du partage des richesses, qui met en évidence que l’austérité pour tous est un choix politique et non une fatalité, ce qui n’a rien, messieurs les ministres, d’irresponsable ni d’inacceptable.

Le travail de nos collègues députés fut aussi riche d’enseignements politiques. Il a mis en lumière des alliances d’opportunité entre le Gouvernement, les groupes de la droite républicaine et ceux de l’extrême droite, nouées afin d’empêcher davantage de justice fiscale dans notre pays.

agite depuis quelques jours le spectre du 49.3. Formidable idée ! Cet expédient aggraverait encore un peu plus la crise démocratique dans laquelle nous sommes plongés. Pourquoi M. Barnier refuse t il de prendre à bras le corps le sujet de la justice fiscale ?

Mais rassurez vous : dans l’hypothèse où cette motion ne serait pas adoptée, nous sommes prêts, avec les forces de gauche présentes ici au Sénat, à démontrer, article après article, que votre projet est particulièrement inadapté et injuste. Nous serons évidemment force de proposition.

Par exemple, pour résorber une partie du déficit public, vous avez décidé de créer un « fonds de résilience des finances locales » en ponctionnant une partie des budgets locaux à hauteur de 3 milliards d’euros.

Messieurs les ministres, les élus locaux sont épuisés d’assumer des politiques avec lesquelles ils sont en désaccord. Depuis plusieurs années, les communes subissent des pertes de recettes réelles, alors que les dépenses, elles, sont en constante progression.

Les collectivités territoriales et les services publics ne sauraient être la variable d’ajustement de libéraux qui profitent de la crise. J’ajoute que l’effort budgétaire demandé aux collectivités aura deux lourds impacts déjà prévisibles

C’est un autre budget que la gauche sénatoriale veut proposer : un budget qui soit au service de la solidarité nationale et non au profit de quelques uns. Nous refusons de renoncer à la justice sociale et à la justice fiscale. Mes chers collègues, nous vous invitons à voter cette motion tendant

Le scrutin est ouvert.

le ministre de l’économie, le directeur de cabinet du Premier ministre n’est autre que celui qui fut directeur de cabinet de votre prédécesseur, Bruno Le Maire, après avoir été directeur général des finances publiques et directeur de cabinet du ministre des comptes publics. Bref, il s’agit de l’homme qui a préparé tous les budgets depuis 2017. n’enlève rien à la responsabilité politique, car la haute fonction publique est là pour exécuter les ordres des élus et non l’inverse. Mais avouez que l’on est en droit de s’interroger. Je mesure l’inquiétude de nos concitoyens face au dérapage budgétaire, face à la situation économique préoccupante que nous connaissons et face à la crise politique qui nous menace.

La récession de 1993, puis la crise de 2008 avaient plongé le solde public dans des profondeurs proches de celles que nous connaissons aujourd’hui. Chaque fois, le retour du déficit sous la barre des 3 % a pris sept à neuf ans. Ne pouvons nous pas échelonner davantage

il faut les soutenir, si l’on veut amplifier cette métamorphose dont dépendent directement notre compétitivité, notre modèle social et notre souveraineté. C’est vrai pour l’industrie ; c’est vrai aussi pour l’agriculture – je ne vous apprends rien.

S’agit il d’endiguer l’hémorragie de nos dépenses ou de remettre en question nos politiques publiques, ce qui, en quinze jours de travail, serait – avouons le – irréaliste, voire dangereux

Être gestionnaire, en « bon père de famille », ne signifie pas être réactionnaire. Le coup porté aux collectivités locales, la brutalité des coupes budgétaires infligées aux solidarités internationales comme l’affaiblissement des ambitions en matière de recherche et d’innovation trahissent des politiques de recul,

Attaquons nous à la prolifération des autorités administratives indépendantes, des observatoires et autres comités Théodule dépendant de Matignon. Les Français attendent un budget de justice sociale et fiscale

Le budget que nous attendons, c’est aussi un budget d’équité territoriale et d’aménagement du territoire : un budget qui répare les fractures et accompagne toutes les communes. Notre pays

Nous serons donc particulièrement attentifs à l’effort demandé aux collectivités locales. Le budget que nous attendons, c’est encore un budget de progrès : de progrès techniques, scientifiques et écologiques ; de progrès humain, tout simplement, ce progrès auquel les radicaux croient encore.

du défi géopolitique qui est devant nous, alliant nos ambitions de défense et de sécurité à des politiques d’aide au développement susceptibles de faire entendre la voix d’une France crédible et sans arrogance. Mes chers collègues,

non par facilité, mais par responsabilité. La France mérite selon nous une autre copie : celle qui préfère l’audace à la peur, la confiance à la défiance et l’action au conservatisme. Nous allons y travailler ensemble. La grandeur de notre pays se mesure non pas à l’aune de ses économies, mais à celle de ses ambitions.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec sincérité et gravité que je m’exprime devant vous.

Permettez moi de penser aux 7 500 ouvriers qui sont aujourd’hui sur la sellette : ceux de Michelin, de Sanofi, de Vencorex, d’ArcelorMittal. Le nombre de fermetures d’usines atteint en effet un seuil inédit depuis la crise de 2008. Or, à nos yeux, 7 500 ouvriers valent mieux que 70 milliards de dividendes. Nous pensons également aux conducteurs de bus de la RATP, aux cheminots et aux travailleurs du fret, à qui on impose une privatisation à marche forcée au nom de la concurrence illibérale et faussée. Nous pensons aux Ultramarins et à la dignité de leur combat face à l’invivable vie chère. Nous pensons aux petits exploitants, éleveurs et agriculteurs, qui ont compris la trahison des traités de libre échange, de l’accord économique Partout dans le pays, jusqu’à la Kanaky, cette multitude de travailleurs, d’agents publics et de familles touchées par la crise du logement a en partage le rejet du libéralisme autoritaire et un intérêt commun au progrès social et écologique. C’est au cœur de cette froide avalanche de plans sociaux et de fermetures annoncées de services publics locaux que nous débattons d’une situation budgétaire totalement inédite. En réponse à cet état que je qualifierais de « désharmonie sociale

Mais nous ne sommes pas dupes, et les citoyens qui nous écoutent doivent avoir conscience de la stratégie de ce gouvernement : laisser le Sénat débattre et arbitrer ensuite les décisions au moyen du 49.3 et de la commission mixte paritaire, cette dernière se substituant au débat de l’Assemblée nationale.

soit les textes les plus antisociaux et réactionnaires que notre pays ait connus de longue date. Le Gouvernement porte la responsabilité de ce coup de force institutionnel. Ce projet de budget s’en prendra aux services publics, aux travailleurs et aux plus vulnérables. Il sous tend de futures réformes structurelles. Malgré quelques évolutions actées côté recettes, le cap reste le même : c’est celui du piège de la dette, qui nous enferme dans une politique fortement récessive et pèsera sur la consommation populaire et les entreprises. J’en viens à la partie recettes. Devant le trouble,

Citons notamment la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), dont les recettes escomptées seraient de 2 milliards d’euros en 2025, en 2026 et en 2027, que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, soit une surtaxe à l’imposition sur les bénéfices, qui ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros

nous assistons à une décentralisation de la dette de l’État. Pourtant, entre 2019 et 2023, l’exécutif a demandé de la transparence et de l’exactitude. Les collectivités ont dégagé un solde cumulé positif de 1,9 milliard d’euros,

au delà des exercices comptables, il est faux d’affirmer qu’assécher les moyens des collectivités permettrait de réduire la dette de l’État, car celles ci ne participent en rien à cet endettement. Il y a un loup, forcément.

raison pour laquelle vous validez le programme d’emprunts de la France sur les marchés financiers, qui atteindra près de 300 milliards d’euros de titres et d’obligations. Je l’affirme, avec Emmanuel Macron, ce sont bien les créanciers de la dette qui ont pris le pouvoir depuis 2017, et le présent budget Monsieur le ministre Armand, vous avez parlé, encore, de transparence et d’exactitude, mais pourquoi ne pas dire que le Haut Conseil des finances publiques estime une nouvelle fois que les prévisions du Gouvernement sont trop optimistes et que la dette augmentera encore ?

du PLFSS, de demander sept heures de travail gratuit aux salariés. La maximisation des profits, grâce à la mondialisation, le marché mondial du travail, le dogme de la concurrence libre et non faussée et l’individualisme libéral sont

nous ouvrons le débat sur le projet de loi de finances pour 2025 dans un contexte politique des plus singuliers, et alors que l’avenir du gouvernement en place est des plus incertains. Messieurs les ministres, vous qui êtes des soutiens de la première heure du Président de la République,

C’est téméraire, tant les décisions du président Macron et de ses gouvernements successifs lors des deux précédents budgets, adoptés au forceps par 49.3, auront été lourdes de conséquences. Leur refus de présenter un projet de loi de finances rectificative (PLFR) en 2024, malgré les alertes appuyées des parlementaires des deux chambres, et leur manque d’anticipation auront abouti à de mauvaises prévisions et à des surestimations de recettes qui ont mené la France dans cette situation critique de déficit abyssal. les recettes fiscales ont fondu, la dynamique économique n’est pas au rendez vous, la croissance est inévitablement atone et le chômage repart à la hausse.

un comble pour des partisans de l’orthodoxie budgétaire et du strict respect des contraintes du pacte de stabilité et de croissance. Le contexte étant posé, le projet de loi de finances pour 2025 dans sa version initiale, celle qui est examinée au Sénat, est un budget de restriction qui se trompe de cible.

sans même vous soucier de l’effet récessif qu’une telle austérité va entraîner. Dans cette perspective, vous voulez imposer 60 milliards d’euros d’efforts, là où la trajectoire de la Commission européenne, au travers de son pacte de stabilité et de croissance, n’en imposerait que 30 milliards. Pourtant, le Premier ministre ne ménage pas ses efforts et mobilise l’ensemble de son gouvernement pour lutter contre la surtransposition des directives européennes, coupable de susciter trop de normes et trop de contraintes – avouez que cela ne manque pas de piquant. yeux des écologistes, la réalité est que ce budget va achever de faire les poches des collectivités territoriales et de l’écosystème des institutions publiques et parapubliques, lesquelles jouent pourtant un rôle central dans l’investissement public et l’accompagnement des forces vives. Par son refus purement dogmatique de lever de nouvelles recettes sur les hauts patrimoines, le présent texte, qui amplifie les injustices et les inégalités, va hypothéquer notre avenir et les conditions d’habitabilité de notre pays. Commençons par les collectivités territoriales.

collectivités locales ne sont pas plus rassurantes. Ainsi, le rabot de 2 milliards d’euros sur les efforts annoncés, négocié par la droite, est largement insuffisant. Alors que les représentants des communes, des intercommunalités, des départements et des régions le Sénat, pour la première fois de son histoire, sacrifie les collectivités sur l’autel de la doxa libérale ! Messieurs les ministres, l’érosion du lien de confiance entre l’État et les élus locaux ne cesse de s’amplifier. Administrer une collectivité, aujourd’hui, c’est jongler avec des dispositifs qui se créent et se défont, dont les règles sont modifiées ou qui ne répondent pas aux promesses initiales. Ces incertitudes, qui rendent l’exercice de planification budgétaire laborieux, voire périlleux, ne sont pas acceptables. En clair, les collectivités territoriales doivent retrouver leur capacité d’agir. Cela passe par un regain d’autonomie fiscale, condition essentielle pour restaurer le lien démocratique et fiscal entre les communes et leurs habitants, ainsi qu’avec les entreprises. S’attaquer aux collectivités, c’est s’attaquer aux gens qui y vivent et qui y travaillent.

attendre et à reporter, engendrera au contraire, dans l’avenir, des coûts bien plus importants, tout en produisant des effets catastrophiques dès maintenant. Votre budget, messieurs les ministres, va à l’encontre de la nécessaire anticipation. Il ponctionne les crédits alloués aux politiques écologiques rénovation thermique des bâtiments, déploiement des énergies renouvelables, sortie progressive des pesticides, protection de la nature et des terres agricoles contre l’artificialisation des sols, lutte contre la déforestation et développement des transports décarbonés. En outre,

il faut maintenant changer de braquet. Vous héritez de sept ans de politiques fiscales qui ont produit de la mauvaise dette et un accroissement de la concentration des richesses et des inégalités. Mais vous gardez le cap,

Pour nous, écologistes, la justice fiscale relève du bon sens ; elle est un enjeu de maintien de la cohésion sociale. Compte tenu de l’explosion des richesses et du patrimoine des plus riches pendant la crise sanitaire, nous proposons de mettre en œuvre la taxe conçue par l’économiste Gabriel Zucman, visant à taxer à hauteur de 2 % la fraction du patrimoine supérieur

Cette taxe pourrait générer 16 milliards d’euros de recettes fiscales, de quoi financer une partie des coupes budgétaires des collectivités et participer au remboursement de la dette. Nous pensons également que le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), assorti d’un volet climatique, et l’élargissement de la surtaxe Barnier sur les bénéfices des grandes entreprises sont de justes solutions. Pour financer nos priorités – l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, la santé, les politiques de l’emploi, la solidarité, le pouvoir de vivre dignement pour les plus précaires, les services publics de proximité et la transition écologique –, nous proposons des réaffectations de crédits dans les dépenses. Ainsi, la rationalisation des primes à l’embauche d’apprentis peut permettre d’économiser près de 1 milliard d’euros par an. Il faut également reconnecter l’économie aux territoires en rétablissant durablement la CVAE, en augmentant le taux des DMTO et en déplafonnant le taux du versement mobilité, dans un contexte de lourds investissements des collectivités pour l’amélioration des transports du quotidien. De meilleures infrastructures engendrent des gains de productivité, monsieur le ministre Armand ! Vous l’aurez compris,

force est de constater qu’il vous en faut peu pour être fier ! Il faut dire que, après sept années de macronisme, le bilan a de quoi faire rêver : 11 millions de pauvres, un taux de chômage qui culminera à plus de 7 % en fin d’année, un record de défaillances d’entreprises,

C’est donc tout naturellement que de cette faillite économique découle le discrédit politique. Celui ci s’est matérialisé à l’occasion des dernières élections législatives, qui ont mis en déroute l’ancienne majorité présidentielle. Il importe en effet de rappeler que votre présence face à nous aujourd’hui tient de l’anomalie démocratique, tant vous êtes illégitime à présenter un projet de loi de finances devant les Français.

leur vieille recette libérale datée. Elles osent nous donner des leçons de sérieux budgétaire, alors que l’état des finances publiques n’a jamais été aussi grave, hors temps de guerre. ministres, vous êtes illégitimes, car le seul véritable gagnant de ces élections, c’est le front républicain, sur lequel vous vous êtes assis en plaçant votre minorité gouvernementale dans la main de l’extrême droite.

votre gouvernement, en raison de son équation politique, se retrouve dans une situation politique insoluble. Il manquait déjà 5 milliards d’euros dans votre budget quand vous l’avez déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, mais, à mesure que le Premier ministre entend satisfaire vos alliés de circonstance, les mesures d’économie fondent comme neige au soleil. C’est ainsi que le groupe Les Républicains du Sénat ne veut pas entendre parler d’une augmentation des taxes sur l’électricité au delà de leur niveau d’avant crise : cela représente un manque à gagner de 3,4 milliards d’euros.

Quant au groupe Ensemble pour la République de l’Assemblée nationale, il refuse le coup de rabot à 4 milliards d’euros sur les allégements de cotisations patronales. Au total, les exigences des parlementaires du socle commun entraîneraient un manque à gagner de 10,5 milliards d’euros. Votre budget s’apparente à un grand jeu de bricolage : on y déshabille Paul pour habiller Jacques, en fonction de la météo politique du moment. Il est ainsi édifiant de

Maintenant que le décor politique est planté, abordons le présent texte. Tout d’abord, comme à l’accoutumée, les hypothèses macroéconomiques qui y figurent ne sont absolument pas crédibles

Le Président de la République a lui même déclaré, à propos du dérapage du déficit, que le problème n’avait pas trait aux dépenses, mais à de moindres recettes. Par conséquent, nous vous apporterons des solutions afin de faire contribuer plus équitablement tous les Français à l’effort collectif. Nos propositions visent à faire pencher la balance du côté de la justice fiscale, quand votre budget nous promet une véritable régression sociale. J’ai entendu dire, çà et là, que nous exagérions en qualifiant ce PLF de budget d’austérité

alors que les déserts médicaux n’ont jamais été aussi nombreux et que même les zones urbaines désormais sont touchées ? Comment ne pas parler d’austérité quand l’écologie sert encore de variable d’ajustement de vos errements budgétaires – je pense aux budgets de MaPrimeRénov’ et au fonds vert pour les collectivités locales ? De toute évidence, vous faites plus grand cas de la dette budgétaire que vous avez vous même creusée que de la dette écologique que vous laisserez à nos enfants. Face à ce budget inique, nous prenons acte des déclarations du Président de la République : le problème réside dans le manque de recettes et non dans les dépenses. Nos propositions visent donc à combler le déficit que vous avez laissé béant. Afin de rétablir un peu de justice fiscale, après sept années d’iniquité sociale, nous proposerons d’augmenter le

au moment même où le CAC 40 accumule plus de 146 milliards d’euros de bénéfices, dont 36 milliards d’euros de superprofits. Toujours animés par la volonté de trouver de nouvelles recettes, nous proposerons de mettre fin à la pratique de l’arbitrage

sur les dépenses et, plus précisément, sur les divers et dispendieux crédits d’impôt qui minent nos budgets depuis des années. Enfin, messieurs les ministres, nous vous demandons très solennellement de ne pas faire des collectivités locales le bouc émissaire facile de sept ans de gestion erratique. Nous refusons d’emblée toutes les ponctions que vous souhaitez leur faire subir. Rappelons que l’État, qui accuse un déficit de plus de 3 300 milliards d’euros, entend faire la leçon aux élus locaux qui, astreints à la règle d’or, doivent présenter chaque année un budget à l’équilibre. Durant nos débats, nous aurons à cœur d’avancer des propositions dont l’adoption garantirait des marges de manœuvre solides à nos élus locaux, notamment l’indexation de la DGF sur l’inflation ou l’augmentation significative du taux des DMTO

et c’est à l’aune de l’acceptation de nos propositions que nous nous déterminerons. En l’état, nous voterons contre ce projet de

nous entamons le débat le plus important de l’année dans un contexte inédit : absence de majorité à l’Assemblée nationale, absence de consensus dans le pays, absence, en réalité, d’un gouvernement responsable, ballotté dans une coalition des contraires et des ambitieux, incapable de se donner une direction – sa longévité même paraît incertaine, oscillant entre quelques semaines et plusieurs mois. La situation budgétaire est dramatique et tous les constats sont déjà connus : des prévisions de croissance surévaluées, une faillite dans l’évaluation des recettes, un cycle économique qui se retourne, une situation internationale plus que dangereuse. Face à cette réalité, la réponse semble évidente : réaliser des économies. Le Gouvernement prétendait fournir un effort immédiat de 60 milliards d’euros ; le Premier ministre affirmait même une fameuse règle des deux tiers deux tiers d’efforts sur les dépenses publiques, un tiers de recettes nouvelles concentrées sur les grandes entreprises et la revue à la baisse des multiples exemptions de cotisations sociales. Néanmoins, la Cour des comptes a bien montré que ce principe affirmé ne correspondait pas à la réalité du budget,

nous devons aussi miser sur la croissance. Seule une économie productive, créant des emplois et générant de l’activité, peut alléger le poids des efforts budgétaires. À cette obligation, par quoi répondez vous ? Par un budget flou et récessif… Alors même que la récession commence et que les plans sociaux s’égrènent, avec leur cortège de drames et de dépenses publiques nouvelles, vous désintégrez la confiance des ménages et des entreprises. Les investissements des entreprises privées sont pourtant déjà en baisse depuis plusieurs trimestres et il en va de même des investissements immobiliers des ménages. Les collectivités portent 70 % de l’investissement public et nous arrivons en fin de cycle des investissements engagés par les élus, particulièrement municipaux ; pourtant, vous cassez la dynamique en leur imposant des coupes insensées de 5 milliards d’euros, alors même que leurs dépenses sont de plus en plus contraintes, sans possibilité d’agir l’arme des impôts locaux, que les gouvernements précédents ont impitoyablement supprimés.

Vous ne touchez pas au coûteux maquis des opérateurs de l’État, lesquels se partagent, dans la plus grande opacité de gestion comme d’action, un pactole de 80 milliards d’euros. Vous ne touchez pas à la gabegie structurelle de l’aide au développement. Ainsi, nos compatriotes seront heureux de savoir que nous continuons de distribuer des centaines de millions d’euros au Mexique ou à la Chine, qui en ont sans doute grand besoin ! Vous ne touchez pas au scandale entourant le développement inefficace de l’éolien, qui donne lieu, des contrats léonins, à des milliards d’euros de dépenses nouvelles. aucune remise en cause non plus du dogme immigrationniste : vous maintenez les 750 millions d’euros de subventions publiques à 1 350 associations pro migrants, soit, sur dix ans, des subventions multipliées par trois pour un nombre de reconduites à la frontière divisé, nous, nous avons pris nos responsabilités en proposant 25 milliards d’euros d’économies réelles, gagées sur la rationalisation des dépenses publiques, la suppression des comités Théodule coûteux et inefficaces, la fin de délires budgétaires comme le plan Vélo de l’État ou les trop nombreuses aides à la presse. est des finances sociales, dont la chambre haute vient de finir de débattre, au lieu de toucher au tonneau des Danaïdes des aides sociales, dont le produit s’échappe par des frontières ouvertes à tous les vents, le Sénat a voté sept heures de travail gratuit pour financer nos retraites. Mes chers collègues, le maintien de notre système social ne peut passer que par la croissance ; nous voulons une France qui travaille, une France des producteurs, non une France des subventions et des profiteurs. Las ! au lieu d’organiser, comme le propose Marine Le Pen depuis deux ans, un dispositif d’augmentation des salaires par le gel des cotisations sociales, vous augmentez ces dernières, au moment même où la consommation des ménages et la confiance des entreprises sont au plus bas.

Par ailleurs, la contribution de la France à l’Union européenne progresse encore, comme si nous pouvions nous le permettre, alors que notre groupe à l’Assemblée nationale l’avait légitimement supprimée. Une fois de plus, ce budget respire le conformisme des solutions éculées, la douceur endormante du déclin, l’irresponsabilité d’un système qui se refuse à être comptable, si ce n’est coupable, de la situation. Il faut conclure. En ces termes, nous ne pouvons l’approuver et nous attendons la rupture, d’abord gouvernementale, ensuite politique,

Mais qu’attendons nous de l’État ? Quelle doit être sa place dans notre société ? L’État, mes chers collègues, est ce que nous décidons collectivement qu’il soit. Et l’État, c’est avant tout ses missions premières,

et la monnaie. Et l’école ! Des missiles traversaient le ciel européen la semaine dernière, mais certains parlent encore de décaler la loi de programmation militaire qui porte nos dépenses à seulement 2 % du PIB. Nous dépensons 38 milliards d’euros par an dans la politique du logement ; c’est trois fois plus que le budget de la justice. Pour quels résultats, mes chers collègues ? Nous sommes d’accord. Alors qu’il a neigé jeudi dernier dans nos villes et dans nos campagnes, des gens continuent de dormir dans la rue et une crise immobilière nous menace. Nous dépensons deux fois plus en paiement des intérêts de la dette cette année que ce que nous allouons à nos forces de l’ordre pour nous protéger. Le

Il doit aussi penser aux générations futures, en investissant dans la lutte contre le changement climatique et dans la recherche et l’innovation, qui nous permettront de nous maintenir dans la compétition mondiale.

il contraint nos concitoyens dans leur liberté et nos entreprises dans leur capacité d’innovation. Aussi n’avons nous presque plus de marge de manœuvre fiscale pour faire face à la crise budgétaire qui nous menace.

face à la chute imprévue et rapide de nos recettes et pour éviter une crise financière grave, le Gouvernement fait le choix d’une augmentation « exceptionnelle, temporaire et ciblée » – je vous plagie, monsieur le ministre – de la fiscalité sur les ménages les plus aisés et sur les plus grandes entreprises de ce pays. Nous nous y résignons,

maintenant aux dépenses. Comme je l’ai indiqué, les sénateurs du groupe Les Indépendants sont attachés aux dépenses régaliennes ; nous soutiendrons donc l’application complète des lois de programmation des ministères de la défense,

de financer les projets des collectivités locales dans les domaines de la performance environnementale, de l’adaptation au changement climatique et de l’amélioration du cadre de vie. Voilà ce que représente 1 milliard d’euros d’action publique : un an d’initiatives écologiques concrètes.

avait été amorcée avec succès, il faut le dire, par Édouard Philippe lorsqu’il était Premier ministre. Ah bon ? La France avait alors su montrer sa capacité à respecter la règle des 3 %.

Il s’agit non pas de sacrifier tel ou tel service public, mais de nous redonner des marges de manœuvre budgétaires afin de pouvoir décider, le moment venu, de renforcer tel ou tel service public.

est, mes chers collègues, la position du groupe Les Indépendants. Vous l’aurez compris, nous nous attacherons à soutenir loyalement le Gouvernement, en faisant porter l’effort majoritairement sur la diminution des dépenses publiques et, pour une part qui doit être la plus réduite possible,

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, avez vous déjà joué à un jeu de société ? ? Ces jeux nous enseignent quelques impératifs auxquels ce projet de loi de finances mériterait de se conformer. La stabilité, tout d’abord : si vous jouez aux jeux de société, vous savez d’expérience que, sans règles claires et précises, il n’y a pas de jeu.

C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible d’accepter la remise en cause des règles régissant le FCTVA ou encore la modification de la trajectoire du malus auto, alors que les industriels ont adapté leur chaîne de production. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible de reporter l’inscription dans la loi du mécanisme de partage de la production nucléaire qui doit venir remplacer le mécanisme de l’Arenh au 1 janvier 2026. Français, acteurs économiques, collectivités locales, tous ont besoin de sécurité juridique. La lisibilité, ensuite : si vous jouez aux jeux de société, vous savez également qu’il est important que la règle soit simple et intelligible ; la complexifier inutilement conduit à perdre les joueurs. Après la crise de 1958, le général de Gaulle, revenu au pouvoir, forme un gouvernement d’union nationale et se consacre à une tâche de stabilisation aux effets durables

Les chantiers de simplification mis en œuvre depuis plusieurs décennies s’apparentent davantage à des opérations de communication qu’à une réelle ambition transformatrice. À l’illisibilité s’ajoutent la perte de sens et l’absence d’une vision de long terme. Comment convaincre les Français de poursuivre l’électrification des usages quand l’électricité se trouvera demain la source d’énergie la plus taxée à la tonne de CO2 émise ? Au vu de l’évolution des prix toutes charges comprises de l’électricité, la fiscalité de rendement a du sens à court terme ; malheureusement, cette orientation envoie un mauvais message aux consommateurs pour ce qui est de leurs comportements de long terme. Il aurait été plus compréhensible d’appliquer la même règle à toutes les consommations d’énergie. Dans un contexte de baisse des prix de gros, les consommateurs sont appelés à rembourser partiellement l’aide que l’État leur a octroyée pendant la crise. Rappelons ici qu’il y va tout de même de 50 milliards d’euros… Entrevoir la victoire sous le prisme du gain budgétaire ou politique, ce n’est pas gouverner : c’est succomber à la tragédie du moment. Savoir ne pas s’y soumettre est ce qui détermine, à mon sens, le sens de l’État. le souci du nombre : si vous jouez aux jeux de société, vous savez qu’en fonction du nombre de joueurs le jeu sera très différent. Jouer au Cluedo à deux ou à huit ne relève pas tout à fait du même niveau de difficulté… Année après année, nous votons un budget pour la France sans tenir compte du nombre de Français et de la chute très inquiétante de la démographie. Depuis 2010, le recul de la natalité est de 19,8 %. La branche famille est la seule branche déficitaire de la sécurité sociale tout un symbole et, surtout, un mauvais signal. Nous indexons les retraites sans tenir compte de la chute vertigineuse du nombre d’actifs cotisant pour les financer. Le projet de loi de finances pour 2025 est le premier à intégrer l’effet en année pleine de la réforme paramétrique de 2023

Nous votons un PLFSS sans tenir compte du vieillissement de la population et des milliards d’euros nécessaires pour financer la dépendance et le grand âge. Comment repensons nous l’organisation de l’enseignement afin d’éviter que n’augmente le coût par élève sans contrepartie quant à l’amélioration du niveau scolaire ? Aux dames, aux échecs, dans tous les jeux de stratégie, si l’on veut avoir une chance de gagner, il faut anticiper les actions futures au moment de déplacer sa pièce. Comme dans les jeux de société, en économie ouverte, il faut tenir compte du nombre de joueurs et anticiper leurs stratégies. l’égalité entre les joueurs. Si vous avez déjà joué au Monopoly, vous savez que la fiscalité n’est pas absente du jeu : deux cases du plateau prévoient un impôt sur le revenu et une taxe ; des cartes dites « Chance » et « Caisse de communauté » peuvent également imposer une contribution particulière. Or ces taxes sont prévisibles et fixes de prélèvement sur bénéfices exceptionnels surgissant au milieu du jeu. Dans notre histoire récente, que fait l’État quand il manque de trésorerie et que les recettes sont moindres que prévu ? Il lève des impôts supplémentaires, ce qui crée de l’incertitude. Ce faisant, il profite de ses prérogatives pour dévier des règles qui s’appliquent à tous. La lecture du dernier baromètre d’Ernst & Young sur l’attractivité est sans appel : en quelques mois, la confiance des investisseurs s’est évanouie. Les incertitudes législatives et réglementaires, ou encore la difficulté à bâtir des plans d’affaires fiables, sont la première cause du report des décisions d’investissement. Pis, les entreprises quittent la France. Tikehau Capital, un fonds d’investissement qui gère plus de 50 milliards d’euros être coté à Wall Street ; le groupe Canal+ va s’introduire en bourse à Londres ; après sept ans d’absence des marchés financiers, Havas sera coté à Amsterdam à partir de décembre.

n’est acceptable que lorsqu’elle permet de corriger ou d’inciter à un comportement plus vertueux. Il y a du sens à punir celui qui ne respecte pas la règle, ou celui qui préfère utiliser un mode de production polluant plutôt que son alternative alternative décarbonée plus onéreuse : c’est une application du principe de liberté et de responsabilité. Très bien ! Au Monopoly, la banque ne fait jamais faillite, elle peut mettre en circulation autant d’argent que nécessaire sous forme de reconnaissance de dette écrite sur du papier ordinaire. Cela fait rêver, messieurs les ministres ! Malheureusement, nos règles financières sont un peu plus complexes et l’État ne

Messieurs les ministres, mes chers collègues, durant les deux prochaines semaines, je crains que nous n’ayons pas le temps de jouer aux jeux de société. Cependant, gardons à l’esprit tout au long de nos débats quelques grands principes : disposer d’une ligne de conduite claire et intelligible ne pas changer la règle du jeu quand celle ci a été intégrée par les acteurs économiques ; anticiper les évolutions démographiques et macroéconomiques pour construire une trajectoire soutenable à long terme doter d’une fiscalité prévisible visant à orienter les comportements ; s’interdire toute politique de l’argent magique. Telles sont, messieurs les ministres, les règles du jeu du groupe Les Républicains. La France mérite que ce gouvernement réussisse. Pour ce faire, il importe de lier le courage à la responsabilité, la rigueur à la créativité, le souci du temps long à celui du plus grand nombre. Une fois ce budget adapté et voté

Monsieur le président,

et trouver la voie des compromis qui nous permettront de sortir de cette crise par le haut. L’objectif premier de ce projet de loi de finances pour 2025 est naturellement le redressement des comptes de la Nation.

et faire face aux nouvelles menaces. Si nous voulons ne pas être acculés par le poids de la dette, qui sera bientôt le premier budget de l’État, si nous voulons garder des marges de manœuvre budgétaires pour faire face aux prochaines crises, si nous voulons continuer à peser en Europe et dans le monde et conserver notre crédibilité,

L’effort sera très important, et même inédit, puisqu’il est chiffré à 60 milliards d’euros. La répartition choisie est de deux tiers pour les dépenses et d’un tiers pour les recettes,

Permettez moi de revenir un instant sur l’effort demandé aux collectivités locales, mes chers collègues. Le groupe RDPI salue le choix du Premier ministre d’un discours de vérité sur la situation particulièrement difficile des collectivités. leurs dépenses incompressibles augmentent, on exige d’elles une participation importante au redressement de nos finances publiques. La semaine dernière, à l’occasion du congrès des maires, nous avons accueilli près de 8 000 élus locaux

La prévision de croissance pour 2025 sur laquelle le Gouvernement a bâti son budget est prudente. Elle s’établit à 1,1 %, soit en dessous des prévisions de l’OCDE et du Fonds La baisse des taux d’intérêt, conjuguée à la baisse de l’inflation, passée sous les 2 %, permettrait de contrebalancer l’effet récessif du choc budgétaire. Près de la moitié des rentrées fiscales supplémentaires de 2025 seraient liées à de nouvelles mesures.

Nous pensons également que l’une des manières les plus efficaces de trouver des recettes est de lutter mieux et plus efficacement contre la fraude et les fraudeurs. Nous présenterons à cet égard une mesure simple de lutte contre la fraude à la TVA : l’interdiction des logiciels de comptabilité dits permissifs autocertifiés.

concerne les dépenses, les objectifs seront certainement plus difficiles à atteindre. En volume, elles devraient légèrement diminuer, pour s’établir à 56,4 % du PIB, soit une baisse de 0,4 Les lettres plafond, qui ont donné le ton de ce PLF, ont pu susciter quelques inquiétudes. Nous estimons qu’il est nécessaire de faire des économies tout en veillant à ne pas casser les dynamiques de rattrapage engagées dans bon nombre de domaines.

elles présentent l’intérêt de prévenir la tentation de faire porter les économies budgétaires sur des domaines que la Nation a jugés comme étant prioritaires et pour lesquels une continuité dans les investissements est indispensable.

ou encore abonder le fonds vert afin de le rapprocher de son niveau actuel. Je ne saurais conclure sans évoquer l’outre mer, où les crises se succèdent. En un an, la Nouvelle Calédonie, en raison d’une crise politique et sociale, et la Martinique, à cause de la vie chère, ont connu troubles et violences

afin que chaque groupe puisse se retrouver dans le texte final. Il n’est pas trop tard ! J’en appelle donc à votre sens des responsabilités, mes chers collègues. Soyons les acteurs d’un compromis, faisons honneur au Parlement et au bicamérisme

L’année dernière, nous avions fait plusieurs propositions pour accroître les recettes de l’État. Si la plupart d’entre elles avaient été adoptées par le Sénat, elles n’avaient pas résisté à l’épreuve du 49.3.

par une plus juste progressivité de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les dividendes distribués étant passés de 30 milliards à 70 milliards

représentent parfois 50 %, voire davantage, de l’ensemble de leurs recettes fiscales. Nous proposerons donc que cette exonération soit justement compensée aux collectivités territoriales et justement indexée.

Faut il en rire ou se morfondre ? Telle est la question. La dette publique a atteint 3 300 milliards d’euros, soit plus de 113 % de notre PIB, un niveau historique qui fragilise notre souveraineté, notre crédibilité sur la scène internationale, mais surtout notre capacité à investir afin de répondre à la complexité des problèmes contemporains qui nous attendent.

suppression de l’impôt sur la fortune, suppression drastique de la taxe d’habitation, disparition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sans oublier la contribution à l’audiovisuel public. plus de 60 milliards d’euros se sont évaporés chaque année depuis 2017. Ce sont précisément ces mêmes 60 milliards d’euros que vous cherchez aujourd’hui désespérément afin de ramener notre déficit sous la barre des 5 % du PIB d’ici à 2027.

Face à une telle situation, comment prétendre financer la transition écologique ou redresser nos comptes publics ? Vos choix budgétaires traduisent une impuissance coupable, aggravée par une obsession comptable déconnectée des réalités sociales et économiques.

de nos collectivités. Les économies et les recettes sont à chercher ailleurs ! Un budget de justice fiscale et sociale est la seule voie crédible pour retrouver une trajectoire budgétaire soutenable tout en respectant les priorités sociales et écologiques de notre pays. En l’état, le texte que vous nous proposez en est très éloigné, messieurs

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames les

vous remercier publiquement, messieurs les ministres, car il répond à l’intérêt général et à ce que demandent nos concitoyens. Ce changement concerne d’ailleurs non seulement les relations avec les collectivités locales, mais toutes les politiques publiques, et donc l’ensemble de ce PLF

si nous ne voulons pas désespérer les Français et faire basculer la France dans une tutelle qui imposerait une austérité d’une tout autre ampleur. Ceux qui ont dirigé notre pays surendetté n’ont jamais remis de l’ordre dans les comptes de l’État ni revu son niveau de dépenses. Il n’est pas question, pour remédier à leurs errements, de mettre inconsidérément à contribution les Français, les entreprises et les collectivités territoriales. Pour autant, il faudra que chacun contribue à un effort socialement et territorialement Le gouvernement actuel a découvert cette situation insoutenable et a dû proposer, dans l’extrême urgence, et dans un cadre inédit, des solutions qui ne sont pas toujours satisfaisantes, mais qui marquent une inflexion que nous allons encore renforcer tout au long du débat qui s’ouvre,

L’alourdissement historique de la dette de l’État, qui atteint 3 300 milliards d’euros, est un fléau qui doit concentrer tous nos efforts. Par delà le stock, c’est la charge de la dette qui inquiète : le flux s’aggrave, en effet, du fait cumulé de son coût et de son volume. En l’absence de redressement appuyé des finances publiques, la charge de la dette de l’État est appelée à doubler d’ici à 2029, et ainsi à approcher la barre folle des 100 milliards d’euros.

alors que l’urgence est de redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux, de réformer l’État pour le recentrer sur le régalien, de mettre fin à l’enchevêtrement des compétences et de faire valoir le principe de subsidiarité ascendante. Les vraies économies sont celles qui simplifient, débureaucratisent et libèrent l’action. Oui, la performance est proportionnelle à la liberté et à la responsabilité. Il faut donc en finir avec la mise sous tutelle et avec l’infantilisation. Il faut, dès aujourd’hui, même dans l’urgence, montrer une voie nouvelle et répondre à la promesse du partenariat avec les territoires et de la décentralisation de la France.

refuser toute mesure rétroactive, donc supprimer l’ensemble de la disposition relative à la remise en cause du FCTVA. Il convient aussi de limiter et d’encadrer les mesures qui touchent les départements dont la situation financière est la plus fragile.

Nous jugerons d’ici à la fin de nos travaux de la manière dont nous aurons été entendus, mais nous attendons d’ores et déjà des signes forts. J’en viens à quelques mots de conclusion. Le pire serait que tout cela ne serve à rien que notre pays, fin décembre, se retrouve dans le chaos plutôt que de commencer à sortir de l’impasse. Mais je veux rester optimiste et continuer de croire que la raison pourra l’emporter. La copie issue du Sénat doit le permettre avant que l’Assemblée nationale ne puisse le confirmer. Si tel n’était pas le cas, notre pays plongerait dans le chaos et verrait le coût de sa dette encore augmenter, ce qui nous précipiterait plus certainement encore vers une mise sous tutelle. La conséquence en serait une situation synonyme non plus de rigueur, mais d’austérité, dont les plus fragiles seraient les premières victimes. La voie du sursaut est possible ; commençons à l’emprunter dès aujourd’hui. La parole

parvenir à voter un budget ? Oui, bien sûr. Le scénario d’un rejet du PLF, et celui du vote d’une motion de censure, est pour moi à écarter absolument. Il n’apporterait rien à la situation de nos finances publiques – rien de positif en tout cas – et occasionnerait de graves difficultés pour nos compatriotes.

très haute. Il faudra rapidement voter un PLFR et se caler sur des prévisions ajustées. Pour aller plus loin, en effet, nous devrons enclencher des réformes structurelles qui ne pouvaient trouver place dans un PLF confectionné en si peu de temps.

Cette politique de l’offre reste une nécessité et souffre sans doute de ne pas avoir été suffisamment financée par des économies équivalentes. Ne l’oublions pas : si notre taux d’emploi rejoint celui de l’Allemagne, alors nos finances seront à l’équilibre.

En cela, les discussions autour du financement des collectivités locales, comme le débat sur l’excès de taxation dans le secteur aérien, seront importantes. Gare à ne pas détruire l’investissement et l’emploi ! Maintenons la vie, les dessertes et les conditions du développement économique dans nos il est urgent de faire des choix dans les missions de l’État et dans le financement des retraites, afin de viser la préservation du niveau de vie des jeunes générations. Une façon d’y parvenir peut être de financer une part de nos retraites et de notre protection sociale par le biais d’une fraction de TVA ou de CSG.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, après les records de chaleur de 2022 et 2023, l’année 2024 est en passe de détenir

prenait enfin conscience de l’enjeu existentiel de la transition écologique. Cet espoir a pris fin avec ce budget, qui acte

ne relève plus de l’austérité : elle signifie le sacrifice pur et simple de toutes nos ambitions en matière de transition écologique. Tous les domaines sont concernés, de la rénovation thermique des bâtiments au soutien aux collectivités territoriales, territoriales, en passant par la biodiversité. Cette trajectoire est très inquiétante ; elle va à rebours de toutes les recommandations des experts. La France a besoin d’un plan d’investissement dans des infrastructures de transport durables. Nous ne pourrons pas remplacer intégralement le parc automobile thermique par un parc électrique équivalent. Il faut donc anticiper et planifier le report vers d’autres moyens de transport.

Des solutions existent pour promouvoir le transport écologique de nouvelles recettes fiscales qui seraient sans impact sur l’activité ni sur les plus précaires la taxation des yachts et des jets privés, le durcissement du malus écologique pour les SUV, l’encadrement des niches fiscales polluantes. Sur tous ces sujets, nous vous ferons des propositions. La France doit également opérer sa transition énergétique en accélérant son soutien aux énergies renouvelables. Or vous amputez le fonds Chaleur, qui accompagne la production de chaleur renouvelable dans les collectivités, de 300 millions d’euros.

Alors que l’Insee a établi, dans l’édition 2024 de son ouvrage, publiée jeudi dernier, que la fin du bouclier inflation avait pesé plus fortement sur les plus modestes, vous aggravez le risque de non recours et de précarité énergétique des ménages. Par ailleurs, alors que la décarbonation passe par l’électrification, le relèvement de l’accise sur l’électricité prévue dans le PLF aurait une fois encore pesé sur les ménages et envoyé un mauvais signal. Nous avons proposé

Alors que la protection de la biodiversité est un objectif essentiel pour l’adaptation au changement climatique, il est prévu que les crédits de la stratégie nationale biodiversité soient divisés par deux.

Ce budget manque d’ailleurs cruellement d’ambition pour ce qui est de lutter à la source contre les pollutions persistantes qui mettent en danger la santé des humains et des écosystèmes. Enfin, vous renoncez à mettre en place le principe pollueur payeur qui évite de reporter les coûts sur la collectivité. Là encore, nous vous ferons des propositions pour réduire les pollutions à la source. Votre coalition a plongé le pays dans la crise budgétaire. Avec ce texte, elle choisit de sacrifier les transitions écologique et énergétique. Ce budget est un budget de renoncement écologique. La parole

Disons le clairement : nous allons examiner un budget difficile, exigeant et qui ne fait plaisir à personne, car il exige des efforts inédits. Il n’est plus possible de se défausser les uns sur les autres, comme l’ont fait récemment certains responsables politiques. Inutile de revenir sur leur attentisme : les conclusions de la mission d’information sénatoriale sur la dégradation des finances publiques depuis 2023 sont édifiantes. Le 15 octobre dernier, la délégation aux entreprises du Sénat a reçu les trois organisations patronales représentatives, ainsi que le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti) : tous les patrons, je peux vous le dire, ont bien conscience de cette responsabilité Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, énième report de la suppression de la CVAE, réduction des exonérations de charges dans le cadre du PLFSS, diminution des aides à l’apprentissage, etc. le coup est dur pour les entreprises, qui sont déjà considérablement fragilisées par une concurrence accrue. À cela s’ajoutent le coût de la surcomplexité normative et l’augmentation des charges incompressibles, telles que le prix de l’énergie ou des assurances. l’ai dit, le discours des dirigeants d’entreprise est celui de la responsabilité face à la dette abyssale de la France. En revanche, ils expriment une crainte : celle que ces mesures exceptionnelles ne finissent par devenir permanentes. Je partage pleinement cette inquiétude. Monsieur le ministre de l’économie, vous avez réaffirmé, ce matin encore, leur caractère provisoire. Nous prenons acte de cet engagement et le Sénat veillera à ce qu’il soit tenu, car le risque pour nos entreprises est immense : nous pourrions entrer dans une récession grave qui serait fatidique pour l’économie française. Nous sommes sur une ligne de crête. Quelque 49 % des investisseurs étrangers ont décidé de réduire leurs projets d’investissement en France.

Cette tendance se renforcera si les baisses des dépenses à destination des entreprises sont reconduites pour les prochaines années. Comme l’ont rappelé les organisations patronales, « le transitoire qui dure, on connaît ! ». La perspective de faillites devrait tous nous alerter. En effet, si le nombre de procédures collectives continue de s’accroître au même rythme que celui qui a été observé depuis le 1 janvier 2024, on peut s’attendre à dépasser les 65 000 procédures sur l’ensemble représentants du Meti lors de leur audition par la délégation aux entreprises, le nombre d’ETI placées en redressement a doublé dans tous les secteurs, de la vente de détail à la construction, en passant par l’aéronautique ou les cosmétiques. Le président du Medef nous a également alertés en pointant la multiplication des procédures collectives, qui concernent tant les petites et moyennes industries que les ETI industrielles. L’emploi doit aussi nous préoccuper. 1 219 suppressions d’emplois par semaine pour les entreprises de moins de dix salariés depuis le début de l’année En trois semaines à peine, il y a autant de suppressions de postes dans les TPE que chez Michelin et Auchan réunis ; et pourtant, personne n’en parle ! Aussi, j’en reviens au principe de responsabilité pour vous rappeler, messieurs les ministres, qu’assume le Gouvernement doit être à la hauteur de ces efforts et des risques qui pèsent sur notre économie. Cela signifie qu’il est urgent de mener des réformes structurelles pour diminuer la dépense publique.

Avançons également en matière de simplification, ce « mal français » si bien documenté par Alain Peyrefitte. L’application du « test PME », tel qu’il a été voté au Sénat, est la seule méthode qui permettra à la France de sortir de sa cage d’acier, afin que l’action publique soit au service de nos concitoyens et de nos entreprises, et non l’inverse. Associons les entreprises aux réformes qui les concernent. Ne reproduisons pas les erreurs du passé je pense par exemple au fiasco du guichet unique, dont les dysfonctionnements graves ont paralysé les entreprises pendant des mois. Messieurs les ministres, mes chers collègues, il nous reste un an d’ici au prochain budget pour diminuer les dépenses publiques. Une fois encore, il faudra faire preuve de responsabilité ! La parole Monsieur le président, messieurs les ministres,

déclenché une polémique. Voilà que nous y sommes bel et bien ; les Français en sont conscients, et il n’est plus possible de repousser les sacrifices nécessaires. Une rapide comparaison européenne permet de mesurer l’état d’urgence budgétaire auquel notre pays est confronté. Notre déficit public – 6,1 % du PIB en 2024 – devrait être le deuxième plus élevé de l’Union européenne, derrière celui

car il marque une rupture dans le sens d’une remise en ordre des comptes publics : il y est procédé à un ajustement équilibré de plus de 50 milliards d’euros qui combine des augmentations de prélèvements obligatoires et des baisses de dépenses. L’heure est enfin venue de nous interroger sur la dépense publique en France, alors qu’elle atteint le niveau le plus élevé de l’OCDE et qu’elle n’a cessé de croître de manière exponentielle ces dernières années.

Pour autant, le financement des missions régaliennes demeure assuré, puisque les trajectoires de financement votées en loi de programmation pour les armées, pour la justice et pour les forces de l’ordre seront respectées. bel et bien de rompre avec la gabegie d’argent public et de tourner définitivement la page du « quoi qu’il en coûte ». La charge fiscale, malheureusement indispensable, demeure mesurée et n’affecte pas les catégories populaires ni les classes moyennes. Dans un pays qui est déjà le plus fiscalisé d’Europe, les marges de manœuvre fiscales sont bien sûr limitées. Mais il nous faut prendre en compte l’impératif de l’urgence. Cette hausse de la fiscalité est nécessaire pour réaliser l’ajustement à court terme.

sont mensongers ou irresponsables. J’ajoute que ce budget sera celui d’un retour à la transparence des finances publiques. Il est tout d’abord fondé sur les hypothèses macroéconomiques du Haut Conseil des finances publiques, ce qui évitera de mauvaises surprises en exécution. Il constitue surtout le point de départ de la reprise d’une trajectoire financière destinée à réduire le déficit public à 5,2 % du PIB en 2025. Je le disais, ce projet de budget n’est pas parfait. Il a bien sûr vocation à être amélioré par les amendements du Sénat. Le Gouvernement peut être assuré non seulement de notre plein soutien dans la voie courageuse qu’il emprunte du rétablissement de nos finances publiques, mais aussi de l’inventivité et de l’expertise du groupe Les Républicains pour corriger ce qui doit l’être. Il est tellement plus facile de promettre le retour de la retraite à 60 ans, de faire des chèques

remercie d’avoir dit que vous ne vouliez pas vous placer dans une démarche d’opposition stérile. J’ai noté que vous étiez membre du parti socialiste ; n’hésitez pas à passer le message